J'ai aussi une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ne siégeront plus parmi nous,

; Désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat, dont je rappelle qu'ils forment le bureau du Sénat ; Proclamation de la constitution du bureau définitif.